Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement. Je souhaite tout d'abord excuser l'absence de M. le président du Sénat, retenu par un déplacement en Ardèche. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook. Au nom du Bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à M. Henri Cabanel, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

le Président de la République a déclaré que celui-ci était « bon à ce stade ». Pourtant, comme l'ensemble des agriculteurs, je m'inquiète du stade d'après. En effet, qu'en sera-t-il demain si cet accord devait s'appliquer en l'état, avec l'importation en provenance des pays d'Amérique du Sud de 99 000 tonnes de boeuf, de 180 000 tonnes de volaille et de 180 000 tonnes de sucre par an ? Comment peut-on demander- à juste raison -à nos agriculteurs d'être plus vertueux dans leurs pratiques et laisser entrer des productions qui recourent massivement aux produits phytosanitaires, comme l'autorise déjà le président Bolsonaro au Brésil ? Le dérèglement climatique fait payer un lourd tribut à nos agriculteurs, avec des phénomènes inédits,

Nos agriculteurs sont fiers de leurs productions, mais ils veulent les mêmes règles que les autres. On ne peut pas en même temps vouloir porter très haut les engagements de l'accord de Paris sur le climat ou défendre un projet de loi Énergie-Climat ambitieux, un accord de libre-échange avec des pays qui, sans scrupule, contribuent à une déforestation responsable de 20 % des émissions de gaz à effet de serre. Cela ne correspond pas à l'attente sociétale. Un bon accord doit être bon pour la France : il ne faut pas sacrifier notre agriculture au profit de notre industrie.

d'obtenir- j'ai même envie de dire « d'arracher » -un certain nombre de mesures propres à rassurer. Je pense en particulier au fait que les quotas qui ont été alloués, par exemple pour la viande bovine,

C'est un non-sens ! Ratifier cet accord revient à sacrifier l'agriculture paysanne au profit de l'agrobusiness mondialisé. Pour garantir une transparence totale, les clauses de sauvegarde ne seront pas suffisantes.

Madame la secrétaire d'État, le 4 novembre 2014, un accord était signé entre le Gouvernement français et l'entreprise General Electric, ou GE. Dans cet accord, GE prenait de nombreux engagements.

Selon les calculs des syndicats de Belfort et de Villeurbanne, qui étaient en visite hier au Sénat, l'entreprise a même supprimé 3 000 emplois.

d'amende que GE a dû verser pour les 1 000 emplois non créés, allez-vous exiger un moratoire sur ce plan social ? Allez-vous engager les poursuites juridiques qui s'imposent pour la non-application de l'accord de 2014 ?

que gérait déjà General Electric au titre de ses turbines à gaz. Je tiens à rappeler que, contrairement à ce que vous avez indiqué, General Electric a recruté 3 000 personnes. Ce n'est que par le jeu des départs naturels

sur un sujet aussi inattendu que celui du lait infantile pour bébés allergiques aux protéines de lait ... Toutefois, la presse se fait l'écho d'une situation assez inédite, et des parents sont plongés dans une véritable angoisse. Il faut savoir nourrissons ne digèrent pas le lait de vache. Cette allergie peut entraîner des symptômes très graves. En revanche, ces mêmes nourrissons acceptent les protéines de riz. Je vous interpelle donc pour évoquer la pénurie de ce lait particulier dont les fabricants connaissent des difficultés d'approvisionnement. L'origine en est identifiée : en janvier dernier, ces produits à base de protéines de riz auraient été infectés par la salmonelle. La production étant ralentie, les usines sont dans l'incapacité de répondre à la demande, qui augmente mécaniquement. Cette pénurie, vous vous en doutez, crée une surenchère des prix. On parle même

Selon l'Association française de pédiatrie ambulatoire, l'allergie aux protéines de lait de vache concernerait de 2 % à 7 % des enfants en bas âge, soit de 16 000 à 56 000 nourrissons- je relève le caractère assez approximatif de ces chiffres Cette situation est doublement problématique : d'une part, en raison des prix anormalement élevés pour les parents ; d'autre part, du fait que certains produits de substitution au lait de riz sont déconseillés par la communauté médicale. Face à Face à l'angoisse, les parents achètent sur internet des produits non validés. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou DGCCRF, et la Direction générale de la santé semblent se renvoyer la balle.

allergiques aux protéines de lait de vache. Environ 1,5 % des enfants de deux mois seraient allergiques aux protéines de lait de vache. Or, comme vous l'avez souligné, en raison de la survenue d'une infection aux salmonelles dans les préparations infantiles du groupe Lactalis groupe Modilac, ces laits ont été retirés du marché par mesure de précaution. Cette situation a entraîné une rupture de stock pour l'ensemble des laits infantiles destinés aux enfants allergiques. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a alerté les professionnels du secteur des aliments de l'enfant, afin de leur faire part de ce problème. La Société française de pédiatrie a établi des recommandations et fourni une liste de produits susceptibles d'offrir des solutions de substitution au lait infantile manquant. Cette liste est disponible sur le site du ministère des solidarités et de la santé. Les parents doivent être vigilants, car certains aliments ne couvrent pas les besoins nutritionnels des enfants, notamment tous les laits végétaux à base de soja, de riz ou encore d'amande, dont on parle parfois et qui sont abusivement présentés comme du lait. abusivement présentés comme du lait. Ces boissons peuvent entraîner des carences nutritionnelles et des manifestations pathologiques. Nous ne les conseillons pas. Afin de trouver le produit adéquat, je demande aux parents de prendre conseil auprès de leur médecin, de leur pédiatre ou de leur pharmacien, qui leur indiquera ce qui convient le mieux à leur bébé.

auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Vendredi dernier, le Président de la République saluait la conclusion de l'accord politique trouvé entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Depuis lors, face à l'unanimité des voix qui s'élèvent pour

Gouvernement à ne pas accepter une demande du Mercosur portant sur un volume d'exportation de viande bovine qui ne serait pas absorbable par le marché européen. La consommation française s'élève à 1,5 million de tonnes équivalent carcasses ; celle de l'Union européenne à 7 millions

La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour le groupe Union Centriste. finances et rejoint en partie celles d'Henri Cabanel et de Daniel Gremillet. Aujourd'hui, des agriculteurs, des parlementaires et des ONG dénoncent les importations déloyales auxquelles les agricultures française et européenne sont confrontées. Depuis 2000, les importations ont presque doublé en France. Or de 10 % à 25 % des produits importés ne respecteraient pas les normes imposées aux producteurs français. La lutte contre ces importations prédatrices constitue un enjeu à la fois économique, de sécurité sanitaire et de santé publique.

Pour garantir l'application de cet article, les représentants des agriculteurs vous ont proposé la création d'un comité composé de la DGCCRF, de la DGAL, de l'Anses et des organisations professionnelles. Allez-vous donner une suite favorable à cette demande ?

commercial est bénéfique pour tous les pays signataires, le monde agricole, les éleveurs et les consommateurs sont inquiets, car l'Union européenne va libéraliser une grande partie de ses importations. Quelles garanties pouvons-nous avoir, que les gros volumes de viande ou d'autres produits agricoles importés soient exempts de produits phytosanitaires ou de molécules interdites en Europe ? La parole est à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances.

D'ici à l'entrée en vigueur de l'accord, le règlement vétérinaire- récemment révisé -de l'Union européenne devrait s'appliquer. À ce titre, en 2022, les importations de viande issue d'animaux ayant reçu des antibiotiques comme activateurs de croissance ou des antibiotiques critiques seront interdites.

à 8 000 kilomètres de Paris, sur une terre guyanaise qui porte les exploits européens de la conquête spatiale, c'est un drame glaçant, récurrent et indigne d'un pays développé qui se joue. En effet, depuis le début des années 2000, la population amérindienne est touchée par une série dramatique de suicides.

Le plus souvent, ces actes suicidaires sont le fait de jeunes adolescents, parfois même d'enfants, pour qui la mort devient l'ultime solution à un mal-être et à un désarroi profonds. Ils sont Wayampis, Wayanas, Tékos, ou encore Kali'na, Palikur et Arawack, tous Amérindiens et Français. Pour eux, le taux de suicide est huit à dix fois supérieur à la moyenne nationale. Notre responsabilité est de dire que cette situation insupportable doit cesser. Vous le savez, madame la ministre, l'appel que je lance aujourd'hui n'est pas le premier. de 2015, un rapport parlementaire proposait déjà trente-sept recommandations pour lutter contre ce phénomène. Force est néanmoins de constater que peu d'entre elles ont été suivies d'effets. En filigrane, nous le savons, c'est la question de la reconnaissance des droits des peuples autochtones- notamment de la ratification de la convention 169 de 1'OIT -qui est posée. Elle est en effet un préalable à la reconnaissance de leur identité et à la restauration de l'estime de soi.

accompagnée d'un psychologue, pour identifier les dysfonctionnements et y remédier, notamment dans ce collège, et accompagner la communauté éducative, qui en a grand besoin. Depuis deux ans, l'État a envoyé des équipes spécialisées pour renforcer le pôle santé dédié à ces questions.

vous le savez, les changements sociétaux qui bouleversent profondément et très rapidement la société amérindienne sont très certainement à l'origine d'une partie de ces gestes de désespoir. En ce qui concerne la convention 169 de l'Organisation internationale du travail, vous savez que notre droit

de l'économie et des finances. La restructuration du service des finances publiques que vous mettez actuellement en oeuvre soulève des inquiétudes auprès des élus locaux, malgré les annonces d'augmentation du nombre de points d'accueil. de points d'accueil. Derrière la promesse de non-fermeture au 1 janvier 2020, on assiste à une disparition des missions de perception, qui sont le coeur des compétences des trésoreries. Dans mon département, pas moins de treize trésoreries sont concernées, alors même qu'elles sont sollicitées par plus de 60 000 usagers chaque année. Oui, madame la secrétaire d'État, il faut prendre en compte les récentes évolutions fiscales, telles que la suppression de la taxe d'habitation ou l'imposition à la source. Toutefois, les trésoreries et la fonction de percepteur gardent une importance capitale. Outre le souci de sécurité que causera le déplacement des usagers, qui devront parcourir de longues distances, la réduction du réseau des trésoreries viendra affecter directement les collectivités et les régies publiques. nous avons des interrogations : si nous saluons la création de points de contact supplémentaires, nous doutons de leur pérennité à moyen et long termes. Nous nous interrogeons aussi sur le rôle et l'utilité de ces futurs conseillers aux collectivités, déployés sur les intercommunalités.

Les élus de nos territoires ne sont pas dans une attitude conservatrice et ne souhaitent pas forcément le. Ils entendent bien formuler des propositions pour garantir un maillage équilibré des trésoreries dans nos départements. Aussi, madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous garantir que les propositions des élus seront étudiées et prises en compte dans cette réorganisation des trésoreries ? Pouvez-vous aussi nous préciser le rôle de ces futurs conseillers aux collectivités ? La parole

Depuis des années, le réseau de la DGFiP- l'un des plus importants de notre territoire avec près de 3 600 points de contact -se transforme pour s'adapter à la fois aux évolutions démographiques et aux changements de pratique. Chaque année, de nombreuses trésoreries étaient ainsi fermées, sans visibilité territoriale d'ensemble et sans que les élus, la population ou les agents soient toujours bien informés en amont. Conscient de l'évolution des missions de la DGFiP- prélèvement à la source, suppression de la taxe d'habitation, etc. -et surtout de la nécessité de s'adapter aux besoins des usagers, le ministre de l'action et des comptes publics a souhaité rompre avec cette pratique en proposant une véritable démarche de concertation, département par département, visant non pas à réduire la présence de ces services publics sur nos territoires, mais, au contraire, à l'accroître de 30 %. Ainsi, madame la sénatrice, il est proposé que cinq communes deviennent de nouveaux lieux d'accueil dans votre département : Sarp, Aureilhan, Bordères-sur-l'Échez, Juillan et Barbazan-Debat. et Barbazan-Debat. Soyez assurée qu'aucune trésorerie n'a vocation à fermer au 1 janvier prochain, bien au contraire. Cette démarche s'appuie sur deux constats auxquels le nouveau réseau de proximité des finances publiques a vocation à répondre part, ces dernières années, les services ont été concentrés dans les métropoles, sans tenir compte des besoins du territoire ; d'autre part, l'implantation des emplois publics doit continuer de jouer un rôle d'amortisseur des inégalités territoriales. Il faut donc prendre en compte les besoins spécifiques liés, par exemple, aux caractéristiques à la fois physiques du territoire et sociales de sa population. Concrètement, les quatre prochains mois seront pour les élus, les agents des finances publiques, les usagers et les représentants de l'État dans votre département l'occasion de débattre, donc d'accueillir vos propositions

interpeller. Nos agriculteurs, qui doivent respecter des normes toujours plus strictes, sont très inquiets de la concurrence déloyale générée par cet accord, qui est en totale opposition avec nos ambitions agroécologiques. Eh oui ! Il s'agit d'une aberration pour notre agriculture, malgré vos dires. Comment pouvons-nous imaginer faire face à l'importation de milliers de tonnes de viande de boeuf, de porc, de volaille et de sucre sans dégâts sur nos filières ? C'est aussi une aberration pour la santé de nos concitoyens. Comment pouvons-nous nous assurer du respect de nos normes face aux pratiques agricoles de ces pays-

écologique et politique. Peut-on ouvrir nos frontières économiques au Brésil, dont le gouvernement fait fi des accords de Paris, déforeste à tout-va et piétine les droits sociaux ? ? Monsieur le secrétaire d'État, nous attendons de vous d'autres garanties que celles que vous venez d'énumérer dans vos réponses et qui sont notoirement insuffisantes pour s'assurer du respect des normes sociales, environnementales et sanitaires et sauver notre agriculture et le climat.

outre extrêmement rentable. Pourquoi a-t-il été supprimé ? Par ailleurs, quelque 1,3 million de Français de l'étranger sont des retraités, expatriés la plupart du temps pour raisons économiques. Permettez-moi d'évoquer ici la véritable persécution administrative que subissent nos compatriotes Français de l'étranger retraités en matière de certificats de vie. Chaque année, ils doivent se présenter aux autorités pour valider leurs certificats de vie, puis les envoyer à leurs caisses de retraite.

Certains retraités doivent effectuer plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre au poste diplomatique français le plus proche ; d'autres n'ont pas les moyens de s'y rendre et voient le paiement de leur retraite suspendu, avec toutes les conséquences que cela implique. Depuis quelques jours, les élus nous ont alertés sur le fait que les consulats ont reçu des instructions leur demandant de ne plus effectuer les validations et de renvoyer les retraités vers les autorités locales. ce cas, ils doivent produire des documents traduits et acquitter une redevance. En outre, les administrations locales peuvent refuser cet acte, en particulier lorsqu'il existe dans le pays une représentation française.

pouvez-vous vous engager sur des délais concrets en matière de mutualisation et de dématérialisation ? Avez-vous clairement informé nos compatriotes retraités et leurs élus de ces nouvelles contraintes ? Accepteriez-vous de donner des instructions aux postes diplomatiques, afin qu'ils puissent accomplir ces missions essentielles pour nos compatriotes établis hors de France ?

une réponse avec une qualité de service identique. C'est le cas au Québec, où une convention est en train d'être élaborée. C'est également le cas en Chine, où la convention est en cours de négociation. Nous sommes en train de diffuser ce modèle partout dans le monde. Là encore,

Voilà quelques années, la SNCF scandait haut et fort qu'elle allait nous « faire préférer le train ». Les trois cents passagers présents à bord du Paris-Clermont du 27 juin dernier ont sans doute une opinion bien différente Bien entendu, nous ne pouvons occulter les circonstances exceptionnelles- conditions météorologiques caniculaires et accident de personne -ayant conduit à la perturbation du trafic. Nous connaissons les problèmes d'entretien du réseau ferroviaire, résultat de décennies de sous-investissement, et nous savons les efforts financiers considérables à entreprendre. Nous sommes tous en mesure de comprendre les cas de force majeure, les aléas climatiques et les accidents. Pourtant, c'est bien une mauvaise gestion de crise qui provoque l'incompréhension et la colère des « naufragés du rail ». C'est sur ce point que le groupe ferroviaire doit revoir ses procédures. À chaque incident, c'est la même rengaine : les dirigeants de la SNCF sont convoqués, ils demandent un rapport, émettent des recommandations. Pour ne citer qu'un exemple, le 23 novembre 2017, il a été répondu à une question écrite de ma collègue Françoise Gatel, à la suite des incidents de la gare de Paris-Montparnasse, de la manière suivante SNCF Réseau a établi un rapport qui a relevé un certain nombre de dysfonctionnements, notamment dans la gestion de la situation et des usagers, et qui comporte neuf recommandations portant en particulier sur l'amélioration de l'information et de la prise en charge des voyageurs. Un an et demi plus tard, ce rapport ne semble pas avoir été suivi d'effets ! Pour compléter ce triste constat, un vent de panique souffle depuis ce matin autour de l'accès aux guichets dans les gares, avec des attentes parfois supérieures à une heure. À quelques heures d'une grande vague de départs en vacances, nombre de nos concitoyens ayant fait le choix vertueux du ferroviaire, j'aimerais connaître, madame la ministre, vos arguments pour qu'ils continuent de préférer le train. La parole

vous avez rappelé les circonstances climatiques exceptionnelles de la semaine dernière. En effet, certains incidents auraient pu être mieux gérés. Je voudrais aussi dire la mobilisation totale des cheminots

Je voudrais aussi souligner leur mobilisation exceptionnelle pour gérer les conséquences des intempéries de ces derniers jours. La fiabilité de nos trains, que ce soit pour les grands départs ou au quotidien, repose tout d'abord sur la remise à niveau de notre réseau. Vous le savez, c'est notre priorité numéro un. Nous allons investir comme jamais, à hauteur de 3,6 milliards d'euros par an pendant dix ans.

tandis que les panneaux d'affichage dépendent de SNCF Mobilités et que les réseaux électriques sont partagés entre les deux entités. Il y aura maintenant une seule entité et un vrai chef de gare. Enfin, je puis vous garantir que nous mettons, depuis deux ans, toute la pression sur la SNCF pour que la fiabilité, la régularité et l'information aux voyageurs soient au coeur de ses priorités. C'est bien le sens de la transformation qu'elle mène. Les premiers résultats sont là : sur les cinq premiers mois de 2019, la ponctualité a progressé de 4,6 points. En outre, depuis les grandes pannes de la gare de Montparnasse en 2017, la SNCF a revu, à ma demande, ses plans de gestion de crise, pour ne plus revivre de telles situations. Madame la sénatrice, les Français comptent beaucoup sur le train. Vous savez notre détermination à ce qu'ils aient un service à la hauteur de leurs attentes. La parole

mutation. La parole est à M. Serge Babary, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la ministre du travail. Avec la réforme de la formation professionnelle et celle de l'assurance chômage, la réforme de l'apprentissage constitue le deuxième chantier social du quinquennat, après celui des ordonnances réformant le code du travail. La « révolution copernicienne », voulue par Mme Pénicaud, s'est traduite, le 5 septembre 2018, par la promulgation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le financement des centres de formation des apprentis, les CFA, a été profondément modifié, en faveur d'un système annoncé comme « plus simple, plus transparent, plus incitatif », avec un engagement ministériel prometteur : « Tout contrat en alternance est financé : chaque jeune et chaque entreprise qui signent un contrat en alternance ont la garantie de bénéficier d'un financement ». Les centres de formation sont ainsi désormais financés au contrat. Si ce nouveau mode de financement, appelé « coût-contrat », est applicable aux contrats d'apprentissage conclus au titre de l'année 2019-2020 par les acteurs privés, nouveaux entrants sur le marché de l'apprentissage, tel n'est pas le cas pour les contrats conclus par les CFA des chambres des métiers et de l'artisanat au dernier semestre 2019. Ces contrats continuent de relever de l'ancien système de financement, appelé « coût préfectoral », avec une compensation de la région dans le cadre de conventions quinquennales. Or cette compensation régionale sera supprimée au 1janvier 2020. À compter de cette date, les contrats conclus au dernier semestre 2019 par les CFA chambre des métiers » ne seront donc plus intégralement financés. Cela concerne quelque 70 000 contrats. Ma question est la suivante : madame la ministre, allez-vous mettre un terme à cette inégalité de traitement ? Un contrat signé à partir de septembre 2019 dans le cadre des conventions quinquennales, non financé par la région à compter du 1janvier 2020, pourra-t-il bénéficier du « coût-contrat » à compter de cette même date ?

De quoi parle-t-on ? D'une réforme ambitieuse que vous avez décrite et qui a été portée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle était fondée sur trois principes très simples : la liberté de créer ou de développer un CFA dans notre pays, en supprimant des obstacles juridiques ou administratifs ; la liberté pour les entreprises d'embaucher des jeunes en apprentissage ; enfin, l'amélioration du statut d'apprenti.

« coût-contrat ». Vous le savez, les chambres de métiers souhaitent une accélération de la mise en oeuvre de la réforme, afin que l'on puisse, entre le mois de septembre et le mois de janvier, répondre à la problématique du financement des contrats qui seraient signés dans cet intervalle.

Nous sommes évidemment en lien étroit avec les chambres de métiers pour discuter de la manière dont nous pourrions accélérer cette mise en oeuvre. Il faut tout de même rappeler deux choses. Tout d'abord, les chambres de métiers peuvent d'ores et déjà bénéficier, dès cette année, du nouveau système de financement pour tous les nouveaux contrats qui sont signés

C'est ce à quoi nous nous engageons, pour faire en sorte que tous les contrats puissent être financés et qu'aucun apprenti ne reste sur le carreau. La parole

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est un phénomène sans précédent qui s'est abattu le week-end dernier sur les départements de l'Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales. Un gros tiers de mon département, soit plusieurs milliers d'hectares, a été touché par des températures supérieures à 45 degrés, avec pour conséquence la destruction totale de parcelles cultivées. La chambre d'agriculture tente d'analyser le phénomène, qui a conduit nos vignes à être comme brûlées au chalumeau.

Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés pour accompagner les exploitants en difficulté. Il s'agit notamment du recours à l'activité partielle pour les salariés, du dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti pour les parcelles touchées,

aux citoyens fortement touchés par cet épisode de canicule, de même qu'aux agriculteurs et aux éleveurs ayant subi d'importantes pertes. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation se rendra demain dans l'Hérault pour mener une réunion sur ce sujet. Il pourra apporter des éclairages sur les mesures immédiates qui peuvent être mises en oeuvre pour accompagner les agriculteurs dans ces difficultés. Ces événements sont exceptionnels ; j'étais moi-même sur place vendredi dernier, et j'ai pu mesurer la température sur le terrain. Vous posez aussi, plus largement, la question de l'adaptation de notre agriculture au changement climatique, car ce qui est aujourd'hui exceptionnel semble devoir se répéter, et il faut mettre en place des outils de gestion des risques. Les événements extrêmes comme la canicule ou les tempêtes de grêle grêle deviendront de plus en plus fréquents. Face à cette situation, il est important que les agriculteurs aient accès à des outils de gestion des risques performants et adaptés aux besoins des filières. C'est pourquoi le ministre de l'agriculture a souhaité lancer une réflexion d'ampleur sur ce sujet, avec l'ensemble des acteurs : agriculteurs, assureurs et financeurs. La première réunion aura lieu au mois de juillet. Il souhaite que ce travail aboutisse d'ici à la fin de l'année 2019. Cette réflexion doit aussi nourrir les discussions en cours sur la prochaine politique agricole commune, tant à l'échelon européen que dans sa déclinaison nationale. Comme vous le savez, les échanges ont déjà commencé. Plus généralement, ces changements climatiques demanderont aux agriculteurs d'adapter leurs pratiques, comme l'ont souligné vos collègues sénateurs dans leur rapport récent. Il faut désormais installer une vraie culture de la prévention. C'est aussi l'objectif de la transition agroécologique que porte le Gouvernement, notamment dans le cadre du groupe de travail « Agriculture » du pacte productif 2025. Nous en Mes chers collègues, j'ai le grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation de membres du Bundesrat conduite par M. Volker Wissing, ministre d'État, ministre pour l'économie, les transports, l'agriculture et la viticulture du Land de Rhénanie-Palatinat, vice-président du groupe d'amitié Allemagne-France du Bundesrat. La délégation est reçue au Sénat aujourd'hui et demain par le groupe d'amitié France-Allemagne, présidé par notre collègue Catherine Troendlé. Il s'agit cette année de la vingtième session de travail commune entre les groupes d'amitié du Sénat et du Bundesrat, qui se rencontrent chaque année, alternativement en France et en Allemagne. La réunion de cette année est structurée autour d'échanges de vues sur deux thèmes : la mise en oeuvre du traité d'Aix-la-Chapelle, d'une part, et l'énergie et le climat, d'autre part. Les rencontres régulières des groupes d'amitié du Sénat et du Bundesrat ont ainsi contribué à créer, au cours des deux dernières décennies, des liens étroits entre nos deux institutions. Ceux-ci ont été confortés par la signature, le 19 mars dernier, d'une déclaration commune entre le Sénat et le Bundesrat, qui s'inscrivait dans le cadre de la nouvelle orientation donnée à la coopération franco-allemande par le traité d'Aix-la-Chapelle. Par cette déclaration, nous avons réaffirmé, avec M. Daniel Günther, président du Bundesrat, notre volonté commune de donner un nouvel élan à la relation franco-allemande et de renforcer la coopération et les échanges entre le Sénat La présence au Sénat de la délégation du Bundesrat aujourd'hui s'inscrit pleinement dans le cadre de ces engagements. Nous sommes particulièrement sensibles à cette visite, qui nous permet de renouveler la profonde amitié qui lie nos deux pays, ainsi que l'étroite coopération entre nos institutions. Au nom du Sénat de la République, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue.